eux ne portait pas de casque. À eux seuls, les cyclistes représentent 2,7 % de la circulation et 7 % des décès. La sécurité routière a évalué la gravité des blessures pour 100 cyclistes, en créant un ratio de gravité. Pour les cyclistes ne portant pas de casque, ce ratio est de 2,3, contre 1,6 pour ceux qui sont coiffés d'un casque. La différence demeure importante. Partant Partant de ce postulat, nul ne peut rester indifférent au risque que nous laissons courir à tous ceux qui ne portent pas le casque à vélo au-delà de 12 ans- comme vous le savez, il est obligatoire avant cet âge ainsi qu'à tous les usagers d'engins à assistance électrique, qui sont totalement exclus du champ d'application de l'obligation, même avant 12 ans. En effet, limiter le port du casque aux seuls utilisateurs de cycles, ce serait ignorer le danger que font courir les nouveaux moyens de transport alternatifs. L'essor des nouvelles mobilités, comme toute nouveauté, entraîne des risques certains. Chacun d'entre nous a déjà été confronté à une situation dangereuse liée à une trottinette électrique. C'est d'autant plus vrai que le développement massif du libre-service pour ces appareils ne promeut que le plaisir et l'intérêt de ce mode de déplacement sans en évoquer les dangers, notamment ceux qui sont liés à la vitesse et à une forme d'instabilité. Ces engins électriques, dont la vitesse peut largement dépasser les 30 kilomètres par heure lorsqu'ils ne sont pas bridés, ne font l'objet d'aucune réglementation quant au port du casque, alors qu'un scooter circulant à une allure similaire y est contraint.

Plus encore, une étude australienne de 2016, qui se fonde sur quarante études internationales, conclut que le port du casque à vélo est associé à une réduction de 51 %, en moyenne, des risques de blessures à la tête et au visage.

blessés au niveau de la tête. On peut légitimement imaginer la protection qu'apporterait le casque s'il était porté par tous les cyclistes, usagers de gyropodes et usagers de trottinettes, en rappelant que la précédente étude évoque une réduction de 50 % des blessures à la tête et au visage. Les chiffres parlent, et rien que les chiffres, auxquels chacun donne une importance particulière pour justifier ses choix. Si des raisons juridiques, plus précisément constitutionnelles, empêchent à juste titre le Parlement d'agir directement et véritablement pour traiter traiter le problème, la commission des lois, je n'en doute pas, partage l'objectif de renforcer la sécurité des usagers vulnérables. En l'espèce, s'agissant du domaine réglementaire, il vous appartient, madame la ministre, d'assumer vos responsabilités sur ce sujet et d'agir en conscience. Certes, vous avancerez la courbe positive et volontaire du port du casque à vélo pour nous indiquer qu'il vaudrait mieux que chacun soit libre de prendre sa propre décision et que le temps fera le travail.

sommes tous conscients du danger, pourquoi protéger uniquement les moins de 12 ans ? Le danger s'arrête-t-il vraiment quand on atteint 12 ans ? Pourquoi ne pas protéger tous les mineurs et, au-delà, tous nos compatriotes ? Pourquoi les athlètes du Tour de France, modèles pour nombre d'entre nous, portent-ils un casque en circulant en moyenne aux alentours de 40 kilomètres par heure, alors que certains engins à assistance électrique permettent aisément d'atteindre cette vitesse, voire de la dépasser ?

à assistance électrique notamment, en le rendant obligatoire. Cela ne découle d'aucune évidence, puisque la compétence s'agissant du port du casque relève du domaine réglementaire. C'est pourquoi j'ai souhaité exploiter un élément du domaine législatif pour présenter cette proposition de loi. Elle s'appuie sur l'article R. 431-1 du code de la route pour créer une infraction de non-port du casque, sur la base de la même infraction à moto.

a pris en compte cette mesure de protection à l'égard de la personne elle-même, sans craindre la diminution de l'utilisation de la voiture pour le secteur automobile. Aujourd'hui, nous nous devons de raisonner pour la protection du plus grand nombre, avec une certaine idée de l'intérêt général chevillée au corps. Le développement des circulations douces ne cessera pas ; les ruptures de stocks régulières sur les ventes de cycles le montrent bien. Domaine réglementaire ou législatif, la visée finale reste la même : agir pour protéger et pour sauver des vies. Cette proposition même s'il eût été bon de mener une action législative immédiate, doit porter le sujet pour l'avenir, en incitant à une sensibilisation plus forte, mais surtout à l'action.

Avant de conclure, permettez-moi de citer Winston Churchill : « On ne devrait jamais tourner le dos à un danger pour tenter de le fuir. Si vous le faites, vous le multiplierez par deux. Mais si vous l'affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduirez de moitié. » En agissant, je suis convaincu que nous protégerons et sauverons des vies. Mes chers collègues, si juridiquement cette proposition de loi peut poser certaines difficultés, car tel est le cas, c'est dans l'action que nous devons nous inscrire pour sensibiliser, protéger et sauver. La parole

et, d'autre part, pour les usagers d'engins de déplacement personnel motorisés, ou EDPM, notamment les trottinettes électriques ou les gyroroues. Je tiens tout d'abord à remercier François Bonneau de nos échanges constructifs. Le port du casque n'est à ce jour imposé qu'aux conducteurs et passagers de vélos de moins de 12 ans, ainsi qu'à tous les utilisateurs d'EDPM, lorsqu'ils sont autorisés par l'autorité de police à circuler hors agglomération. L'infraction à cette obligation est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Comme vous l'avez dit, cher collègue, il existe un consensus scientifique sur l'efficacité du casque en cas d'accident protège des traumatismes crâniens ou de la fracture du crâne, même si son efficacité décroît au-delà d'une certaine vitesse, à 45 kilomètres par heure, voire à 30 kilomètres par heure. Les professeurs de médecine ou de biomécanique que nous avons entendus ont plaidé pour le port du casque obligatoire, s'appuyant notamment sur l'étude d'une université australienne selon laquelle le port du casque à vélo est associé à une réduction de 51 %, en moyenne, des risques de blessures à la tête. Quant à l'utilisateur non casqué d'un EDPM, il risque, selon les travaux de l'université de Strasbourg, une fracture du crâne dans près de 95 % des cas et une commotion cérébrale dans 90 % des cas, lorsque la vitesse dépasse les 20 kilomètres par heure. Pourtant,

Or la mortalité cycliste a augmenté de 21 % depuis 2010 et le nombre de blessés en EDPM de 40 % en un an. La proposition de loi de François Bonneau nous invite donc à passer de l'incitation à l'obligation.

tout d'abord d'étendre aux cycles et aux EDPM la possibilité d'immobiliser ou de mettre en fourrière un véhicule, telle qu'elle existe déjà pour les deux-roues à moteur, en cas de défaut du port du casque ou de gants. Elle prévoit, ensuite, de sanctionner l'infraction de l'usage sans casque de ces véhicules, par l'amende déjà applicable dans la même situation aux deux-roues à moteur. Bien qu'elle partage l'objectif de renforcer la sécurité des usagers de la route vulnérables, la commission des lois n'a pu que constater que ce texte relevait de la responsabilité du Gouvernement. En effet, l'obligation du port du casque est une disposition de nature réglementaire, tout comme les peines applicables aux infractions contraventionnelles. De surcroît, la commission a estimé que l'immobilisation ou la mise en fourrière d'un vélo ou d'un EDPM pouvait être disproportionnée et source de difficultés pratiques dans sa mise en oeuvre par les forces de l'ordre. En revanche, le débat est légitime sur cette importante question de sécurité routière et de santé publique. Les nombreuses études scientifiques sur le sujet attestent la protection qu'offre le port du casque en cas d'accident à vélo ou à bord d'un EDPM. Il est donc crucial de l'encourager fortement. S'agissant du vélo, nous avons estimé qu'il fallait trouver un équilibre entre volontarisme et prudence, compte tenu de l'intérêt du port du casque, d'une part, et du risque de décourager la pratique, d'autre part. La Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) s'y oppose, pour ce motif Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous propose de ne pas adopter cette proposition de loi. Sans me tromper de débat ni confondre le port du masque avec le port du casque, je considère qu'il vaut mieux convaincre que contraindre. En outre, comme je l'ai expliqué,

comme texte d'appel, pour interpeller le Gouvernement sur ses ambitions en matière de sécurité routière. Madame la ministre, comment comptez-vous encourager le port du casque à vélo ? Envisagez-vous de généraliser l'obligation du port du casque pour les engins de déplacement personnel motorisés ?

Pour conclure, je veux remercier une nouvelle fois François Bonneau de la qualité de sa démarche et de l'intérêt des interrogations qu'il nous soumet. Je remercie également par avance Mme la ministre de la qualité des réponses qu'elle voudra bien apporter aux questions que nous nous posons tous.

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, dès l'automne 2017, les Assises nationales de la mobilité ont montré l'importance de donner toute leur place aux mobilités actives, notamment au vélo, dans les politiques mises Pour faire évoluer la situation, le Gouvernement a d'ailleurs décidé d'engager, dès le 14 septembre 2018, un plan Vélo qui porte l'ambition de faire du vélo un mode de transport à part entière. massif, mais cohérent et précis, ce plan vise à tripler la part du vélo dans nos déplacements quotidiens d'ici à 2024. Son lancement a permis de lancer une nouvelle dynamique, qui repose sur la mobilisation de tous les acteurs de terrain, collectivités, entreprises et associations. Récemment, le député Guillaume Gouffier-Cha a été chargé d'une mission parlementaire sur l'industrie du vélo en France. Ce plan est accompagné d'un volet qui vise la sécurisation des itinéraires cyclables le renforcement des mesures de sécurité routière en faveur des cyclistes, car le manque de sécurité est l'un des principaux freins au développement de ce mode de déplacement. Pour cela, le Gouvernement a créé le fonds national Mobilités actives, doté de 350 millions d'euros, pour soutenir, accélérer et amplifier les projets de création d'axes cyclables structurants dans les collectivités. Je suis très heureuse de pouvoir vous annoncer que 533 projets ont été financés dans ce cadre. Pour accompagner la hausse de la part des cyclistes dans le flux des véhicules et pour renforcer leur sécurité, le Gouvernement, sous l'impulsion de Gérald Darmanin, ministre de l'intérieur, a adopté une approche globale et mis en oeuvre des actions très diversifiées pour améliorer encore la sécurité des cyclistes. Nous avons notamment engagé des mesures législatives et réglementaires, des mesures éducatives et nombre de campagnes de communication. Comme vous le savez, les dix dernières années ont été marquées par des évolutions du code de la route en faveur des mobilités actives, et notre gouvernement s'engage fortement en ce sens. Le plan Vélo a poursuivi cette dynamique par la création du principe de prudence à l'égard de l'usager vulnérable, qui se concrétise dans l'article R. 412-6 du code de la route. De plus, la redéfinition de certaines zones de circulation apaisée incluant des zones piétonnes et des zones 30 lorsque celles-ci sont pertinentes localement doit se faire, toujours en concertation avec les habitants. Par ailleurs, la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a introduit l'obligation pour tous les véhicules lourds d'apposer un autocollant matérialisant leurs angles morts, pour mieux les indiquer aux usagers vulnérables qui circulent à proximité. Cette obligation simple et peu coûteuse, qui est rapidement opérationnelle, résulte d'un amendement parlementaire que je veux saluer. Nous déployons également de nombreuses mesures éducatives, notamment la mesure n°

La sécurité à vélo est aussi une affaire d'information des usagers. C'est en ce sens que, sous l'impulsion du ministre de l'intérieur, la Délégation à la sécurité routière porte régulièrement des campagnes d'information et de communication spécifiques aux risques liés à la pratique du vélo, plus particulièrement à l'équipement des cyclistes et à leur visibilité. En 2020, nous avons accompagné la sortie du confinement de plusieurs actions de communication, menées sur le terrain, puis nous avons porté, dès l'automne, une large campagne concernant le port des équipements de sécurité et l'amélioration de la visibilité des cyclistes. lancé une autre campagne sur les mêmes thèmes au printemps 2021. Il est important de préciser que seuls les vélos et les deux-roues motorisés bénéficient de campagnes spécifiques. Vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement agit en matière de sécurité à vélo. En ce qui concerne la proposition de loi que vous examinez aujourd'hui et qui vise, très légitimement, à renforcer la sécurité des usagers du vélo et des engins de déplacement personnels motorisés, je ne puis que saluer l'intention l'intention de M. le sénateur François Bonneau, auteur de ce texte, que je remercie chaleureusement de porter ce sujet dans le débat public. Cette proposition de loi prévoit la modification du code de la route pour sanctionner l'infraction de l'usage de vélos et d'engins de déplacement personnel motorisés sans casque, par l'amende déjà applicable, dans la même situation, aux deux-roues motorisés. Elle vise également à permettre l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule conduit dans ces conditions, ou en cas de non-utilisation des autres équipements de sécurité obligatoires. Toutefois, l'immobilisation et la mise en fourrière des cycles ou des trottinettes se heurtent à de nombreuses difficultés pratiques, qui rendent ce mode d'action assez peu opérationnel, et même parfois impossible. Du fait de la nature de ces engins et de leur mode de gestion, de nombreuses interrogations surgissent quant à la procédure à mettre en oeuvre, qu'il s'agisse des conditions d'immobilisation, d'immobilisation, de l'enlèvement et du stockage en fourrière, des modalités de notification, de l'expertise et de la mise en destruction, le cas échéant, ou bien encore du montant et du paiement des frais de fourrière. En outre, à la différence des véhicules immatriculés, aucun moyen de contrainte, tel que la confiscation du certificat d'immatriculation ou l'inscription de l'immobilisation au sein d'un système d'immatriculation des véhicules, ne paraît à ce stade pouvoir dissuader l'usager de reprendre son véhicule en l'absence des forces de l'ordre. Concernant l'obligation du port du casque, s'il existe un consensus scientifique sur le fait que le casque, à condition qu'il soit bien conçu, adapté et porté, réduit de manière importante le risque de fracture crânienne ou de lésions neurologiques, force est de constater que, à l'échelle internationale,

la Nouvelle-Zélande et certains États des États-Unis. En l'état actuel du droit, le port d'un casque homologué et attaché est obligatoire uniquement pour les enfants de moins de 12 ans, qu'ils soient passagers ou passagers ou conducteurs d'un cycle, sous peine d'une contravention de quatrième classe. Par ailleurs, selon l'observatoire des comportements de la sécurité routière, lors de l'introduction de cette obligation, en 2016, dans les grandes agglomérations,

Enfin, comme le montrent les statistiques, sans réglementation contraignante, le port du casque à vélo chez les plus de 12 ans est en constante progression. C'est dû, d'une part, au principe de l'enfant prescripteur- il s'agit de donner l'exemple pour convaincre ses enfants -, et, d'autre part, au caractère très efficace des campagnes de communication destinées à faire progresser l'usage du casque

madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi entend répondre à une préoccupation bien légitime,

De fait, la France connaît une croissance de l'accidentologie cycliste, alors que celle de l'automobile diminue. Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, la mortalité cycliste a augmenté de 27 % entre 2010 et 2019, contre une diminution de la mortalité routière en général de l'année 2019, quelque 187 cyclistes ont perdu la vie dans un accident de la route, tandis que plus de 1 600 autres ont été hospitalisés. Dès lors, le port du casque apparaît comme étant le moyen le plus sûr de protéger sa tête en cas de collision ou de chute. Les traumatismes crâniens sont nombreux, et les blessures dues à un choc au niveau de la tête représentent la première cause de décès chez les cyclistes. À ce jour, bien qu'il soit uniquement obligatoire pour les cyclistes et les passagers de moins de 12 ans, en vertu de l'article R. 431-1-3 du code de la route,

proposition de loi de notre excellent collègue François Bonneau nous offre l'occasion d'attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de mieux protéger cyclistes et utilisateurs des nouveaux moyens de micromobilité. À titre personnel, je saisis aussi l'occasion, dans le cadre de cette discussion générale, de vous alerter, madame la ministre, au sujet d'autres moyens de transport pour lesquels des améliorations pourraient être envisagées en matière de sécurité. Je pense notamment aux quads, car mon département est rural. En effet, une meilleure sécurisation pourrait être apportée à leurs utilisateurs. Ces engins sont souvent utilisés dans les exploitations agricoles, afin de surveiller les troupeaux et les clôtures, ou encore pour contrôler l'état des cultures. Ils sont aussi utilisés de manière ludique. Très utiles et pratiques en milieu rural, ils sont malheureusement, chaque année, à l'origine de nombreux accidents, principalement dus à leur retournement.

Bonneau, il ne pourra cependant pas la voter, car l'obligation du port du casque à vélo relève du domaine réglementaire.

tricycle ou quadricycle à moteur depuis 1980, les cyclistes échappent encore à cette obligation. En effet, en l'état du droit, l'obligation du port d'un casque homologué et attaché concerne exclusivement les enfants de moins de 12 ans, qu'ils soient passagers ou conducteurs d'un cycle. Je souscris bien évidemment

Ainsi, les sportifs qui roulent à vélo à une vitesse élevée portent généralement le casque ; les parents, eux, dotent de plus en plus les jeunes enfants de casques. Je reste favorable à une forme de liberté et à une appréciation éclairée du risque pour chaque utilisateur. est d'autant plus essentielle que les Français n'ont jamais eu autant envie de pratiquer le vélo. Cette dynamique est positive pour de nombreux territoires, notamment ruraux, qui bénéficient parfois de ces retombées économiques.

pas pour autant que l'accidentalité à vélo progresse elle aussi, avec son triste lot de blessés et de tués. Quand on interroge ceux qui hésitent- ils sont nombreux -à se mettre au vélo au quotidien, la première raison qu'ils invoquent pour y renoncer, c'est l'insécurité.

mais les données sur l'accidentalité et les analyses des politiques en matière de vélo dans les autres pays nous montrent qu'une telle obligation serait contre-productive. Non seulement elle enrayerait l'essor du vélo et les gains très importants auxquels il conduit en termes de santé publique, mais elle n'aurait

vitesse, les dispositifs anti-angles morts des véhicules lourds- il ne faut pas en rester au seul autocollant -et la généralisation de l'apprentissage du savoir rouler à vélo. Déjà,

Sans abuser des chiffres et des expertises, quatre données significatives sont à prendre en compte. Premièrement, sur les dix dernières années, les cyclistes gravement blessés à la tête correspondent, fort heureusement, à seulement 1,09 % du total des blessés.

l'obligation du port du casque, là où elle a été appliquée, a rendu le vélo moins attractif et a découragé la pratique, annulant ainsi cet effet sécurité par le nombre. Oui, les promoteurs de la présente proposition de loi ont raison de chercher à sécuriser la pratique du vélo, mais la solution qu'ils proposent n'est pas la bonne. Je suis strasbourgeois et je connais les travaux de l'équipe du professeur Willinger de l'université de Strasbourg.

de la sécurité. Un plan Vélo renforcé pour les infrastructures cyclables, une généralisation ambitieuse de l'apprentissage du savoir rouler, la mise en oeuvre d'un système de voirie et de déplacement sûr, les dispositifs anti-angles morts des véhicules lourds, telles sont les politiques publiques pertinentes à déployer

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs années, nous assistons à une recrudescence de la pratique du vélo, des trottinettes électriques, des gyropodes et autres skateboards électriques. Ce phénomène emporte des conséquences en termes de sécurité routière, et l'on sait que la moitié des cyclistes accidentés ne porte pas de casque. La question du port du casque se pose donc à nous toutes et à nous tous, à la société dans son ensemble. En l'état actuel du droit, le port d'un casque homologué et attaché est obligatoire uniquement pour les enfants de moins de 12 ans, passagers ou conducteurs d'un cycle. cycle. L'article unique de la proposition de loi vise à généraliser le port du casque obligatoire à tout conducteur d'un véhicule, que ce dernier soit à moteur ou à assistance électrique.

en se limitant au seul volet répressif, sans être accompagnée d'une campagne de prévention tendant à favoriser l'acceptation du port du casque, la proposition de loi risque de ne pas atteindre pleinement son objectif. Ensuite, ce texte

il conviendrait d'envisager d'autres évolutions législatives et réglementaires, notamment pour favoriser le développement des transports collectifs. Enfin, sur le fond,

l'utilisation du domaine public en autorisant l'implantation de ces véhicules. Toutefois, il est impérieux d'aller plus loin et d'aborder également la régulation des usages sous l'angle de la protection d'un autre utilisateur de la voirie

puisque ces véhicules ont vocation à circuler sur la route, il faut rappeler qu'un effort important doit être consenti pour développer plus encore les pistes cyclables et les voies dédiées aux vélos. Certains départements s'y engagent d'ores et déjà. C'est une nécessité pour sécuriser celles et ceux, toujours plus nombreux, qui ont pu faire le choix de se déplacer à vélo ou en trottinette, par exemple, ces dernières années.

chers collègues, avant tout, je tiens à saluer l'initiative de notre collègue du groupe Union Centriste, François Bonneau, qui nous permet de débattre aujourd'hui d'un texte relatif au port du casque à vélo, parmi d'autres moyens de transport.

de son travail. Tout en partageant la motivation et la sincérité de la démarche sur ce sujet important, il a su faire preuve de pédagogie, en expliquant les difficultés qui seraient rencontrées sur les plans juridique et pratique si ce texte venait à être adopté. Vous l'avez compris, mes chers collègues, ce texte nous invite à passer de l'incitation du port du casque à vélo à l'obligation. Il s'articule autour de deux axes. D'une part, il vise à étendre la possibilité d'immobiliser ou de mettre en fourrière un véhicule à moteur pour les conducteurs de deux-roues à moteur, en cas de défaut du port du casque ou de gants moto, aux cycles et EDPM. Ces sanctions seraient également rendues possibles en cas de défaut du port d'autres équipements obligatoires destinés à la sécurité du conducteur, comme le gilet réfléchissant ou un éclairage complémentaire.

C'est ainsi que, en 2019, sur 187 cyclistes tués et 4 783 cyclistes blessés, la moitié ne portait pas de casque. Mais que faire pour renforcer la sécurité d'usagers vulnérables sur la route ? cela a été rappelé, depuis une loi de 2017, le port du casque à vélo n'est obligatoire que pour les seuls conducteurs et passagers de moins de 12 ans. En ce qui concerne le port du casque chez les personnes majeures, bien que des travaux scientifiques attestent de son efficacité en cas d'accident, cet usage chez les cyclistes est encore minoritaire,

vous le savez, le Sénat est la chambre des territoires, mais il n'est pas la seule institution à les mettre en avant : je pense au Tour de France, cette belle fête populaire et rurale qui rythme nos étés depuis déjà plus d'un siècle

Le Belge Wilfried Nelissen vint percuter un policier légèrement avancé pour prendre une photo, entraînant avec lui Laurent Jalabert. Le champion français souffrira de fractures au niveau du visage, passera plusieurs semaines à l'hôpital et ne remontera sur un vélo qu'au mois d'octobre suivant. Il ne portait pas de casque ! Presque vingt-cinq ans plus tard, le 24 juillet 2018, le Tour traversait le département de la Haute-Garonne. Le Belge Philippe Gilbert courait en tête et s'est engagé dans la descente du col de Portet-d'Aspet. Dans un virage qu'il négocia mal, il fonça sur le parapet et s'envola dans le ravin, faisant une chute de plus de deux mètres. L'image est terrible, particulièrement impressionnante ; elle dissuaderait quelques parents d'inscrire leur enfant dans des écoles de cyclisme ... Toutefois, après un rapide diagnostic, le médecin donna son feu vert, et le coureur reprit la course. Ce n'est peut-être pas la seule explication, mais figurez-vous que, à la différence de Laurent Jalabert, Philippe Gilbert portait un casque. Il faut dire que, entre 1994 et 2018, la réglementation des courses cyclistes a changé, puisque, en 2003, le casque est devenu obligatoire, ce qui avait provoqué de nombreuses réticences à l'époque. on n'envisagerait plus de revenir sur cette décision, qui concerne des cyclistes pourtant professionnels, des sportifs formés et aguerris circulant sur des routes fermées sans autres usagers. Que faudrait-il décider pour protéger nos concitoyens en chemin pour le travail sur leurs bicyclettes, tout aussi pressés, mais peut-être moins adroits que notre champion du monde Julian Alaphilippe, se faufilant entre les voitures, d'un angle mort à un autre ?

une telle obligation relèverait du domaine réglementaire quand nous nous plaignons sans cesse de l'inflation législative. En outre, son application pourrait se montrer particulièrement difficile, voire contre-productive. Il serait difficile de la mettre en oeuvre, car la question de l'immobilisation des véhicules risquerait de créer une surcharge importante de travail

travail. Cher François Bonneau, je souhaiterais louer votre intention de protéger les cyclistes, mais elle apparaît comme une fausse bonne idée et semble même contre-productive du point de vue de l'intérêt général. Tout d'abord, vous créez une sanction sans incrimination, un contrôle et une peine sans qu'un principe proportionné ait été défini en amont. En effet, l'obligation du port du casque figure bien dans l'exposé des motifs, comme l'a souligné le rapporteur, mais pas dans le texte lui-même. De plus, le dispositif est de nature réglementaire et ne concerne pas le législateur, sans compter que la détermination de la peine relève du code pénal. Vous proposez dans un second temps un dispositif

Gouvernement. Cher François Bonneau, vous êtes tout comme moi un cycliste. Vous vous protégez et vous souhaitez encourager la pratique du vélo. Je sais que vous ne voulez pas faire peur aux cyclistes. Vous avez cité Churchill

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le texte dont nous débattons ce matin, déposé par François Bonneau et plusieurs de ses collègues, tend à instaurer une obligation de port du casque pour tous les cyclistes, mais également pour tous les usagers d'engins de déplacement personnel motorisés. L'article unique qui nous est présenté vient également punir l'absence de casque de la même peine d'amende que dans le cas d'une conduite de moto sans casque. L'objectif- mieux protéger les usagers -est partagé sur toutes les travées de notre assemblée. Dans le bilan dressé en 2020 par l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, la gravité d'un accident, établie en calculant le nombre de tués pour 100 blessés, est en effet plus élevée pour les cyclistes ne portant pas de casque que pour les autres : 2,3, contre 1,8 en agglomération ; 19, contre 11 hors agglomération. D'un point de vue normatif, cette proposition de loi fait suite à deux mesures récentes démontrant que les pouvoirs publics se saisissent pleinement de la problématique : une mesure réglementaire de 2017 a rendu le port du casque obligatoire pour les enfants âgés de moins de 12 ans, qu'ils soient conducteurs ou passagers d'un cycle ; une autre mesure, toujours d'ordre réglementaire, a étendu l'obligation, en 2019, aux utilisateurs d'EDPM lorsqu'ils sont autorisés par l'autorité de police à circuler hors agglomération.

l'automne 2020 et au printemps 2021, visant le port des équipements de sécurité et l'amélioration de la visibilité des cyclistes. Sans obligation, donc, le taux d'équipement naturel en casque chez les plus de 12 ans est en constante progression- preuve que les démarches de sensibilisation fonctionnent. En effet, l'objectif doit être de trouver un juste équilibre entre la sécurité et le soutien au développement de ce mode de déplacement, afin de ne pas décourager la pratique collective, en essor depuis maintenant deux ans. Il s'agit d'un enjeu de santé publique et d'un enjeu environnemental. Entre le 1 janvier et le 31 décembre 2021, le nombre de passages de vélos a été de 28 % plus important qu'en 2019. C'est une augmentation notable.

Si mon groupe votera contre le texte, je voudrais saluer cette proposition de François Bonneau, dont nous partageons l'esprit, et reprendre quelques éléments avancés par le rapporteur Jérôme Durain.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs années, nous remarquons une évolution de nos moyens de transport en faveur de la micromobilité : vélos, trottinettes, gyropodes ou skateboards électriques rencontrent un succès croissant. La crise sanitaire a amplifié l'utilisation de ces modes de déplacement. Ainsi, le marché du cycle a augmenté de 25 % de 2019 à 2020, atteignant un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros.

apportent des bienfaits physiques aux utilisateurs, au travers de la pratique du sport. Ils sont bénéfiques à l'environnement, car leur utilisation contribue à la diminution des gaz à effets de serre. D'ailleurs, dans mon département de la Manche, nous nous sommes engagés dans cette politique volontariste d'aménagement et de valorisation des voies cyclables, afin de favoriser les déplacements doux, utilitaires, mais aussi le tourisme de nature et de loisirs. Par l'aménagement des anciennes lignes de chemin de fer ou des chemins de halage, nous avons pu mettre en place des boucles vélos locales sur routes partagées et, ainsi, bénéficier d'un maillage dense de plus de 1 000 kilomètres d'itinéraires cyclables. Beaucoup reste néanmoins à faire. à faire. Le problème de la sécurité de ces engins devient de plus en plus critique. En 2020, sur le plan national, les cyclistes représentaient 6 % de la mortalité routière, cela a déjà été souligné, avec 178 tués, dont la moitié sans casque. Depuis mars 2017, le port d'un casque homologué et attaché est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, qu'ils soient passagers ou conducteurs d'un cycle, et le non-respect de cette obligation est sanctionné par une contravention de quatrième catégorie.

heure. Nous constatons que 86 % des propriétaires d'EDPM portent un casque, ce nombre s'abaissant à 9 %, seulement, pour les engins en libre-service. Le port du casque, même s'il est fortement conseillé, n'est pas obligatoire pour les cyclistes de plus de 12 ans et les adultes. Il est vrai que de nombreux scientifiques attestent de l'efficacité du casque en cas d'accident. Une étude de l'université d'Australie de 2016, regroupant 40 études internationales, conclut que le port du casque réduit de 51 %, en moyenne, les risques de blessures à la tête et au visage. En France, si la mortalité cycliste, stable depuis trois ans, a tout de même augmenté de plus de 21 % depuis 2010, le nombre de blessés en EDPM s'est accru de 40 % en une seule année. Le casque est porté par 31 % des utilisateurs en 2020 selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Si la proposition de loi a pour but de rendre obligatoire le port du casque pour tous les utilisateurs de moyens de micromobilité, on peut noter qu'elle ne fait pas consensus. La Fédération française des usagers de la bicyclette s'y oppose notamment, craignant que cette nouvelle contrainte ne décourage les utilisateurs de la pratique du vélo, dont les bénéfices pour la santé publique sont connus. Malgré tout, ce texte a le mérite de soulever un débat légitime de sécurité routière et de santé publique. Autant étendre le port du casque obligatoire pour les EDPM me semble une mesure de bon sens, autant l'imposer pour les cyclistes me paraît plus complexe. à ce dispositif de sécurité par des campagnes de communication sur le danger du non-port de casque, en particulier dans les établissements scolaires ; renforcer la sécurisation des infrastructures, par exemple en peignant des bandes cyclables sur la chaussée ou en développant le nombre de voies réservées à ces moyens doux de mobilité innover pour rendre le casque moins contraignant : tout cela permettrait une acceptabilité progressive de cet équipement de sécurité, afin de concilier l'effet bénéfique de l'exercice physique permis par la pratique du vélo avec le souci important d'une protection maximale pour les usagers de cycles. laissons les cyclistes adultes prendre leur responsabilité concernant le port du casque ! Cette proposition de loi vise également à étendre la possibilité d'immobiliser ou de mettre en fourrière cycles et EDPM, au titre de l'article L. 431-1 du code de la route qui s'applique actuellement aux deux-roues motorisés, lorsqu'il y a défaut du port des équipements obligatoires- casque et gants -, mais aussi en l'absence de gilet réfléchissant hors agglomération ou de l'éclairage complémentaire pour les EDPM. Ces sanctions sont applicables au conducteur, comme à son passager éventuel. Ces mesures sont d'ordre réglementaire et ne relèvent pas de la compétence du législateur. De plus, la possibilité de mettre en fourrière un véhicule en cas de non-respect du règlement entraînerait des difficultés pratiques- elle nécessiterait la mobilisation d'agents et entraînerait des coûts supplémentaires. Ces mesures de rétorsion seraient également peu efficientes, car, contrairement aux deux-roues motorisés, tels que les motos ou les scooters, ces engins n'ont pas de carte grise, et la mise en oeuvre prévue au 1 mars 2022 semble totalement irréaliste. Le partage de la chaussée par ces différents types de véhicules doit relever du bon sens et du civisme de chacun. Ce serait, je pense, la meilleure des protections.

collègues, je rappelle les termes de l'article 26 du règlement du Sénat : « L'auteur ou le premier signataire d'une proposition de loi ou de résolution peut toujours la retirer, même quand la discussion est ouverte. La proposition de loi relative au port du casque à vélo et dans le cadre d'autres moyens de transport est donc retirée. Mes chers collègues, nous allons maintenant